Quel que soit l'opérateur de transport public employeur- régie directe, société d'économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation -, la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l'accomplissement de l'ensemble de leurs tâches sur les lignes du réseau qui les emploie et uniquement sur celles-ci. Pendant plusieurs dizaines d'années, et jusqu'à récemment, toutes les caisses d'Urssaf avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail au travers d'une doctrine fondée sur le droit social et la réalité d'usage de cette carte. Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constitueraient un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales. Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaître cette carte de service comme une carte nécessaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité. locatif. Quel est l'avis de la commission ? En vertu de l'article 24 de cette convention, certains salariés peuvent se voir attribuer une carte de service qui permet l'utilisation des transports à titre professionnel. Il semble que certaines caisses caisses d'Urssaf auraient considéré que la CSG devait être prélevée sur ces cartes, au motif qu'elles peuvent être également utilisées à des fins professionnelles. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d'inscrire dans la loi que ces cartes de service sont exonérées de CSG. Si, effectivement, ces cartes sont considérées comme des instruments de travail,

vous proposez de modifier le code du tourisme pour rendre obligatoire l'octroi par les employeurs de chèques-vacances à compter de 2021. Un amendement de ce type avait été déposé, sans qu'il soit

une autre méthode, qui en vaut bien d'autres, sachant qu'on peut parfois faire confiance à nos concitoyens, sous le contrôle de l'administration fiscale. Nous prévoyons une valeur locative déclarative, qui permettra de s'adapter aux situations territorialement extrêmement diversifiées

et CIID). Il ne modifie pas l'ajustement et la suppression de certaines conditions de désignation des membres de ces commissions, inscrites à l'article 52 du projet de loi de finances. Mais, compte tenu de la difficulté concrète à mobiliser des commissaires remplissant ces conditions, ces mesures me paraissent bienvenues. Elles témoignent d'ailleurs du dialogue fructueux entre la DGFiP et les associations d'élus. Le présent amendement vise à les compléter. Tout d'abord, en prévoyant de faciliter les conditions de quorum. En effet, actuellement, les commissaires qui acceptent de siéger à la commission communale ou intercommunale des impôts directs et qui ne participent plus aux travaux de la commission ne peuvent être remplacés tant que ceux-ci n'ont pas formalisé leur démission auprès du président de la CCID ou de la CIID, ce qu'ils ne font pas le plus souvent, y compris après relances. De plus, il est proposé de préciser que le président de la CCID puisse choisir, à l'occasion d'une réunion, de se faire représenter par un autre membre élu de la collectivité, qu'il aura spécialement désigné pour cette réunion. En effet, dans les plus grandes collectivités, il est souvent extrêmement compliqué de trouver des disponibilités du maire ou de l'élu aux finances pour la tenue de ces commissions. Il s'agirait donc pour lui de pouvoir mandater, par exemple, l'adjoint chargé des questions d'urbanisme

ainsi libellé : La parole est à M. Yvon Collin. Cet amendement vise à réintroduire les avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) lors de l'évaluation des bases des locaux professionnels. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a en effet modifié les missions des commissions en matière de locaux professionnels : les nouveaux paramètres d'évaluation ne nécessitent plus que les commissions dressent avec le représentant de l'administration fiscale la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives, puisque les tarifs sont mis à jour de manière permanente sur la base des relevés des loyers. Toutefois, la participation des CCID et CIID à l'évaluation des bases des locaux professionnels permettrait aux collectivités locales de mieux prévoir les recettes de la collectivité et contribuerait à la fiabilisation des bases avant leur intégration à la base cadastrale et aux rôles des impôts directs locaux. Grâce à leur connaissance du tissu économique, les commissaires peuvent émettre un avis sur les catégories de locaux choisies par les déclarants ou sur la ventilation des surfaces déclarées, qui a un impact sur le niveau des bases imposées. Les commissaires peuvent également signaler à l'administration fiscale d'éventuelles démarches d'optimisation des déclarants visant à supprimer les mécanismes atténuateurs sur des valeurs locatives en baisse. Enfin, les commissaires peuvent continuer de participer à l'exhaustivité des mises à jour cadastrales eu égard aux autorisations d'urbanisme délivrées par la collectivité. En outre, il est important de veiller au maintien du rôle des commissions communales et intercommunales dans la détermination des bases d'imposition, et ce à la veille de la mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, dont le futur dispositif pourrait être la simple transposition de celui qui a été appliqué pour les locaux professionnels. Ces commissions pourraient donc également ne plus être sollicitées pour apporter leur concours à l'établissement des valeurs locatives des locaux d'habitation. Quel est l'avis de la commission ? Sur le fond, je comprends Quel est l'avis de la commission ? Sur le fond, je comprends l'intérêt de solliciter les élus, au travers des commissions, en cas de désaccord avec l'administration fiscale.

S'agissant de l'association des élus, l'administration fiscale propose une offre de services aux collectivités territoriales dans le cadre d'un partenariat en vue de stabiliser la base fiscale. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusqu'à ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur, ne serait-ce que pour ne pas mettre les élus eux-mêmes en difficulté. Il faut retravailler la relation entre les élus, dont on sait bien qu'une très

d'implantation et le siège social de l'entreprise de distribution, et on assiste à une tendance à la multiplication des grandes surfaces qui semble excessive en comparaison avec d'autres pays européens. Cette tendance semble liée au fait que les nouvelles grandes surfaces soient moins rentables que les anciennes. Pareille situation est révélatrice de problèmes concernant ce secteur. Pour des raisons économiques et de rentrées fiscales, les communes peuvent être tentées d'autoriser des grandes surfaces non ou peu rentables, alors que les régions le seraient peut-être moins : elles

pour étendre la procédure d'abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal. L'article L. 64 A du LPF uniquement une règle d'assiette et n'entraîne pas automatiquement l'application de sanctions fiscales, comme l'a démontré notre rapporteur général dans son rapport n° 147 déposé au cours de la session 2018-2019. Il n'y a pas eu de coordination pour modifier l'article 1729 du code général des impôts : la majoration de 80 % des droits n'est pas applicable au montage à but principalement fiscal, à l'inverse de ce qui est prévu pour les opérations à caractère exclusivement fiscal. Par ailleurs, l'instruction fiscale du 3 juillet 2019 a exclu du champ d'application de l'article L. 64 A du LPF l'impôt sur les sociétés au motif qu'il serait désormais traité exclusivement

fiscale. Élisabeth Lamure et les cosignataires de cet amendement estiment qu'une telle interprétation restrictive aboutit à priver une entreprise de son droit de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, alors qu'elle pourra continuer à le faire si la contestation de l'administration fiscale concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou les compléments de TVA. Par ailleurs, la situation est d'autant plus absurde que, lorsque l'article L. 64 A du LPF entrera en vigueur le 1janvier 2020, les entreprises pourront de nouveau, en matière d'impôt sur les sociétés, saisir le comité de l'abus de droit fiscal. Il existe, en outre, une incertitude juridique sur la situation applicable à l'impôt sur les sociétés pendant l'année 2019.

dire, monsieur le ministre,

Ils veulent également que soient étudiés l'application de la résolution votée par le Conseil de l'Europe ainsi que l'impact financier et fiscal, pour l'État et les collectivités françaises, d'un accord similaire à celui qui prévaut avec le canton de Genève.

pour le seul commerce électronique, le paiement scindé : l'acte de paiement de l'acheteur provoque la perception, à la fois, bien sûr, du prix de vente, mais également de la TVA. C'est actuellement le seul actuellement le seul moyen, avec ce qui a déjà été voté par le Sénat et d'ailleurs repris par le Gouvernement concernant la responsabilité solidaire des plateformes, de s'assurer que la TVA est effectivement payée,

Je remercie le ministre d'avoir envoyé le rapport. Je lis la première page de la synthèse : « Dans un monde où tous les paiements seraient effectués par voie électronique, le paiement scindé " à la source " est probablement une solution moderne. Pour l'heure, il ne pourrait être envisagé que de manière partielle (certaines transactions certains secteurs) ». C'est précisément ce qu'on propose ! Le paiement scindé généralisé n'a pas de sens ; le paiement scindé sur le commerce

Votre article prévoyait simplement la remise d'un rapport : le Gouvernement n'a pas besoin d'un article pour se faire remettre un rapport, il peut en faire autant qu'il veut ! Encore une fois, nous souscrivons à la facturation électronique et au paiement scindé

notre pays s'est toujours fait fort d'être à la pointe de la défense et de la protection des données personnelles lorsqu'elles sont, mes chers collègues, la prolongation de votre vie, de vos choix et de vos idées. En cela, chaque question qui touche aux données personnelles est forcément un sujet de libertés publiques. Autant le dire, je ne suis pas opposé à l'utilisation d'informations provenant des réseaux sociaux pour des enquêtes par les services des douanes ou les services fiscaux. D'ailleurs, ces services le font déjà. En revanche, je m'oppose fermement au principe de l'aspiration massive de données, notamment personnelles, sur les réseaux sociaux et à leur traitement par un logiciel algorithmique en vue de lutter contre la fraude fiscale. Nous passerions alors d'une logique de ciblage à une logique de chalutage.

Dès lors que vous aurez utilisé, mes chers collègues, ces services, l'administration fiscale pourra, avant toute infraction, à tout moment, « aspirer »- le terme est peu élégant, mais assez éclairant -les données personnelles que vous aurez inscrites sur ces plateformes.

pour réaffirmer la souveraineté fiscale et numérique de l'État.

Monsieur le ministre,

pourquoi il nous paraît normal que l'interdiction de recourir à des prestataires externes s'étende non seulement aux opérations de conservation et de traitement des données, mais encore aux opérations de collecte.

2016 a créé un mécanisme de bail réel solidaire (BRS), afin de favoriser des opérations d'accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier, acquis par un organisme de foncier solidaire (OFS), et du bâti, acquis par le ménage. Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict, se développent sur l'ensemble du territoire, avec l'appui d'un certain nombre de collectivités locales. La loi de finances rectificative pour 2016 a permis aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'appliquer un abattement de 30 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) due par les ménages qui acquièrent leurs logements dans ces conditions. Pour encourager davantage de telles opérations, il est proposé de modifier le texte, afin de permettre aux collectivités de porter cet abattement à un niveau supérieur à 30 %.

plusieurs mutations immobilières. Ainsi, dans le cas le plus courant, l'organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti- c'est la première mutation -, puis concède des droits réels, un BRS, à un opérateur- il s'agit de la deuxième mutation -, lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage, ce qui constitue la troisième mutation. Chacune de ces opérations est en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement. La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes, en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la deuxième mutation. Toutefois, contrairement aux schémas existants dans les opérations d'accession classiques, lorsque l'organisme de foncier solidaire achète un terrain, il ne peut pas prendre l'engagement de construire pour diminuer le montant des droits dus sur son acquisition, car ce n'est pas lui qui va construire : c'est un opérateur, avec qui il aura signé un bail réel solidaire. De même, si l'organisme de foncier solidaire achète un logement ancien, il ne pourra pas prendre l'engagement de revendre pour diminuer les droits dus, car il revendra non pas l'immeuble à proprement parler, mais uniquement des droits réels sur le bâti. Ces situations peuvent donc conduire à la perception de droits au taux plein, une première fois lors de l'acquisition réalisée par l'OFS, par l'OFS, puis lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages. Afin d'éviter ces situations et d'encourager de telles opérations, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les OFS au droit fixe de 125 euros, étant entendu que la cession des droits aux ménages reste, quant à elle, soumise aux droits d'enregistrement selon les règles de droit commun, en fonction des modalités du contrat et de l'âge de l'immeuble. Quel est l'avis de la commission

puisqu'il bénéficie du taux réduit de 5,5 % de TVA, lequel est maintenu dans les mêmes conditions dans le cadre de l'article 8 du présent projet de loi de finances, et d'une exonération de la taxe de publicité foncière. Si le Gouvernement ne voit pas d'obstacle au principe d'une exonération facultative, sur délibération des conseils de département,

Favorable.

monsieur le ministre,

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Jeansannetas. L'article 58 vise à créer une réduction d'impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d'un service d'intérêt économique général, dès lors que nombre de ces acteurs ne seront plus éligibles à la réduction d'impôt Madelin. l'initiative revient à mon collègue Joël Labbé, vise à compléter cette mesure, en faisant entrer dans le champ du dispositif les foncières exerçant une activité d'acquisition et de gestion par bail de biens agricoles dans des conditions caractérisant un service d'intérêt économique général, exclues du dispositif dans le texte issu de l'Assemblée nationale et dont l'équilibre économique est donc menacé à très court terme. Son adoption permettrait de protéger les foncières agricoles telles que Terre de liens.

ce qui facilite l'installation de personnes n'ayant pas les moyens d'investir dans l'achat du foncier, leur apporte un accompagnement lors de leur installation et sort des terres agricoles de la spéculation foncière, tout en leur assurant une vocation agricole à long terme. De plus, les baux signés entre Terre de liens et les agriculteurs contiennent des clauses environnementales, permettant d'assurer le respect des ressources naturelles et de la biodiversité. Pour ces acteurs, le plafond de versements éligibles à la réduction d'impôt serait fixé à 15 millions d'euros maximum, soit un montant supérieur à leur collecte collecte actuelle au titre de la réduction d'impôt Madelin et de nature à garantir la pleine compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d'aides d'État.

en élargissant ce mandat aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale. Ainsi, cet amendement vise à protéger toutes les foncières « entreprises solidaires d'utilité sociale » (ESUS), dont l'équilibre économique est menacé à très court terme. La

constituerait une forme de réparation pour les veuves d'anciens combattants. L'amendement

Selon les dispositions actuelles de l'article 195 du code général des impôts, les veuves d'anciens combattants ne peuvent aujourd'hui bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire qu'à une double condition : qu'elles aient plus de 74 ans et que leur conjoint décédé ait pu en bénéficier de son vivant.

supplémentaire de son vivant : il faut simplement qu'il ait perçu sa retraite de combattant de son vivant, c'est-à-dire à partir de 65 ans, voire 60 ans, sous conditions.

prévoit une modification de l'article 195 du CGI afin que la demi-part fiscale soit attribuée, à partir de 74 ans, à toutes les personnes veuves dont le conjoint défunt avait bénéficié de la retraite du combattant ». Si le rapporteur « n'est pas défavorable à cette mesure, il note qu'il subsistera une différence entre les veuves dont le conjoint ancien combattant est décédé après 65 ans (ou 60 ans dans les cas où il remplissait les conditions pour bénéficier de la retraite du combattant à cet âge) et celle dont le conjoint est mort avant de bénéficier de la retraite du combattant ». Le présent amendement vise à assurer l'équité entre toutes les situations,

Cet aménagement se justifie par le fait que les exigences en termes de travaux sont identiques, que le PSMV soit approuvé ou seulement en cours d'étude. Dans un cas comme dans l'autre, la protection des intérieurs des immeubles est assurée, ce qui différencie le PSMV des autres cas de figure pour les sites patrimoniaux remarquables. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement et ce sous-amendement sont conformes aux prescriptions des différents rapports commandés par le Gouvernement. Ils permettent à la fois de stabiliser la dépense fiscale

en adaptant le dispositif concerné aux zones qui connaissent le plus de contraintes en termes de travaux de restauration immobilière, en les faisant bénéficier du taux le plus élevé. Le taux dérogatoire de 30 % se justifie par l'importance des contraintes architecturales résultant de l'application du PSMV pour les investisseurs.

À la différence du dispositif Pinel, la location des locaux ayant bénéficié du Malraux n'est subordonnée à aucun plafond de loyer ni de ressources du locataire. Ainsi, eu égard à l'importance du levier fiscal qui permet de réaliser jusqu'à 120 000 euros de réduction d'impôt sur quatre ans, il apparaîtrait disproportionné que l'investisseur puisse héberger, même dans le cadre d'un contrat de bail, un parent ou un enfant, même non rattaché à son foyer fiscal. Enfin, modifier le pourcentage d'investissement en réduisant la part du foncier devant être acquis

ainsi libellé : La parole est à M. Antoine Lefèvre. L'acquéreur d'un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d'impôt dite « Pinel » que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l'acte authentique d'acquisition. Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître le maître d'ouvrage sous tension pour respecter l'échéance légale. Il présente toutefois deux défauts. Tout d'abord, il méconnaît la réalité des programmes immobiliers à deux égards. D'une part, la réalisation de certains programmes immobiliers, en raison de leur complexité, nécessite plus de trente mois. Cette complexité résulte, par exemple, de leur taille, de leur hauteur, de la présence de carrières, de la nécessité de réaliser des fondations spéciales ... Ces critères concernent en particulier les zones tendues où le dispositif Pinel est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l'artificialisation d'espaces naturels. D'autre part, de nombreux aléas peuvent affecter des programmes immobiliers, indépendamment de leur complexité : prescription de fouilles archéologiques, recours contentieux, faillites d'entreprises du BTP, découverte d'espèces protégées ou de pollutions imprévues, etc. Dans ce cas, le délai de trente mois prive l'acquéreur du bénéfice de la réduction d'impôt pour un motif indépendant de sa volonté, ce qui va à l'encontre de la protection du consommateur. Enfin, ce dispositif ne ménage aucune souplesse. La seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, n'en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités- force majeure, ou recours contentieux. Il paraît donc souhaitable d'assortir ce délai de trente mois d'une forme de souplesse en s'inspirant de ce que prévoit déjà le code général des impôts dans un cas analogue- en l'espèce, le respect d'un engagement de construire dans un délai de quatre qui conditionne le bénéfice d'une exonération de droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière. Dans ce cas, en effet, il est possible de demander aux services fiscaux le bénéfice d'une prolongation de délai pour une période d'un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP. effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d'améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget ». Ce dispositif d'incitation fiscale dans l'ancien, destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu'ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé, n'est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme « coeur de ville ». Cet amendement vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d'une expérimentation, le dispositif d'incitation fiscale dans l'ancien, dit « Denormandie ». La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans. Le dispositif ne serait étendu qu'aux métropoles ayant conclu une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat de type renouvellement urbain.

et, pour chaque commune ou partie de commune éligible, par type de logement, les plafonds de loyers et plafonds de ressources des locataires. Les dispositions de cet amendement nous semblent conduire à un encadrement des pouvoirs du préfet de région dans la fixation des plafonds de loyers et de ressources, puisque celui-ci ne pourra déroger à une disposition mentionnant que le loyer et que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Or il semble au Gouvernement que le maintien de la possibilité de dérogation correspond à l'esprit de cette expérimentation qui doit permettre

vise à mettre en oeuvre. Or les subventions et dispositions fiscales contribuant à endommager ou artificialiser les espaces protégés sont contraires à la mise en oeuvre de ce même plan qui tend à « créer de nouvelles aires protégées et conforter le réseau écologique dans les territoires ». Cet amendement a donc pour objet de supprimer les subventions aux constructions neuves dans certains espaces protégés, tout en maintenant la possibilité d'aides publiques pour la rénovation et la restauration des bâtiments existants à l'intérieur même de ces espaces. Les constructions sans subventions ne sont pas visées. Les régimes Pinel et Censi-Bouvard, le PTZ, l'exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le prêt action logement, les prêts compte épargne logement (CEL) et prêt épargne logement (PEL), la récupération de la TVA sur les résidences de services, ainsi que les exonérations de taxe foncière sur d'impôt sur les sociétés et de TVA sur les logements sociaux sont visés par cet amendement.

au titre de l'acquisition de certains logements- dispositif Censi-Bouvard -, notamment lorsqu'ils sont compris dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code du travail.

intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en étendant le champ du dispositif d'autorisation, qui relève de la compétence des départements, substitué partiellement à l'agrément. Le présent amendement vise à tirer les conséquences, au sein de l'article 199 du code général des impôts, des modifications apportées aux modalités de reconnaissance des services prestataires par la loi ASV.

du Gouvernement ? La réduction d'impôt Censi-Bouvard bénéficie aux personnes qui investissent dans une résidence de service, notamment pour personnes âgées, âgées ou handicapées. Ces établissements doivent avoir obtenu un agrément qualité prévue à l'article L. 7232-1 du code du travail.

et non plus celui de l'agrément. Les auteurs de cet amendement proposent de tenir compte, dans le code général des impôts, des modifications apportées par la loi ASV en y introduisant le régime de l'autorisation pour l'activité d'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à cet amendement

a eu une excellente intuition : le Gouvernement est très favorable à cet amendement qui met en oeuvre une recommandation de la Cour des comptes. Dans son rapport sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme de janvier dernier, la Cour a demandé la désignation d'une administration pour effectuer le contrôle de la contribution forfaitaire sur les contrats d'assurance de biens

Merci